rectifié . Nous proposons que les modifications apportées au champ d'application du taux réduit de la TVA aux livraisons d'immeubles réalisées dans le cadre d'un bail réel solidaire (BRS) s'appliquent également, par mesure de cohérence, aux livraisons à soi-même (LASM) d'immeubles de ce type.

aux livraisons de logements sociaux et aux livraisons à soi-même des mêmes logements pour les organismes de logement social. Il paraît donc pertinent de faire de même dans le cadre des logements destinés à faire l'objet d'un BRS. La commission

Entre 2006 et 2019, le coût du logement a augmenté en moyenne deux fois plus vite en Corse que sur le continent, et le coût du foncier quatre fois plus vite. Pour répondre à cette aggravation des inégalités et de l'exclusion sociale, l'Assemblée de Corse a adopté un nouveau règlement des aides en faveur du logement et de l'habitat le 27 septembre 2019. Cet amendement vise à appliquer la baisse du taux de TVA, de 10 % à 5,5 aux logements locatifs sociaux construits dans la collectivité de Corse, conformément au règlement des aides en faveur du logement et de l'habitat adopté par l'Assemblée de Corse. Ce règlement doit contribuer à ce que la Corse, où l'offre de logement social locatif s'élève à 10 %, rattrape la moyenne nationale, qui s'élève à 17 %. Quel est l'avis de la commission

dans quelle mesure les logements locatifs sociaux réalisés directement par les collectivités territoriales pourraient bénéficier d'un taux réduit de TVA. Quel est

pour les constructions neuves de logements locatifs sociaux aux opérations portant sur des logements anciens, sous les mêmes conditions de financement et de conventionnement que pour les logements neufs. L'article 278 du code général des impôts définit les logements sociaux susceptibles de bénéficier d'un taux réduit de TVA, taux de 5,5 % ou 10 %, ce en fonction du type de logement et du type de ménages auxquels ils sont destinés. Historiquement, l'application de ces taux réduits était prévue uniquement pour les constructions neuves. Toutefois, compte tenu de la raréfaction du foncier dans les zones en tension, où les besoins de logements sociaux sont élevés, de plus en plus d'opérations de logements sociaux sont issues de la transformation d'immeubles anciens déjà bâtis, que les bailleurs sociaux affectent, après travaux de rénovation, au logement social. Le législateur a pris en compte cette situation en admettant, dans certains cas, que les taux réduits de TVA puissent s'appliquer à des opérations réalisées à partir d'immeubles anciens. Il est proposé d'aller plus loin en autorisant, de manière générale, l'application des taux réduits aux créations de logements sociaux réalisées à partir de la transformation d'immeubles anciens, sous les mêmes conditions et garanties que celles qui sont applicables aux constructions neuves. Cette proposition permettra notamment de favoriser les montages dans lesquels une entreprise vendrait un immeuble ancien à usage de bureaux à un bailleur social, en vue de sa transformation

d'un travail de concertation avec les professionnels, qui a débouché sur le pacte d'investissement pour le logement social. Ce pacte privilégie les logements

présenter l'amendement n° I-237. Notre amendement tend à rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l'ensemble des opérations de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux financés en PLAI et PLUS, quel que soit leur lieu d'implantation. La crise du logement abordable doit nous inciter à construire massivement des logements qui répondent aux besoins des Français. La France doit reprendre un rythme soutenu de production de logements abordables et soutenir les familles modestes dans leur projet d'acquisition et de mobilité résidentielle. Comment résorber l'habitat indigne si l'on ne peut pas reloger les familles ? Comment mettre en place le plan Logement d'abord si nous ne disposons pas d'une offre de logements adaptés ? Comment soutenir la production de logements sociaux si nous privons les organismes HLM de leurs ressources ? Comment demander aux maires de mettre en oeuvre les politiques publiques quand ils n'en ont plus les moyens ? Lorsqu'en 2017 nous avons voté au Sénat l'augmentation du taux de TVA de 5,5 % à 10 % pour la construction et la rénovation des logements sociaux,

appliquée par les bailleurs. Depuis le début du quinquennat, le groupe socialiste refuse ces choix politiques, qui répondent à des logiques purement budgétaires. Il est difficile d'accepter que l'effort de réduction budgétaire continue de toucher les plus pauvres ; voilà qui est totalement contradictoire avec la volonté affichée du Gouvernement de demander aux offices HLM de loger encore plus de personnes démunies, notamment dans le cadre du plan Logement d'abord. Le retour à un taux de TVA à 5,5 % est à la fois une urgence et une nécessité pour revenir à un rythme de construction de logements sociaux qui puisse répondre aux besoins des Français. L'amendement

financés en PLAI et PLUS, pour tout lieu d'implantation. Seules les opérations portant sur des logements financés en prêt locatif social (PLS) seraient maintenues au taux de 10 %. Ce dispositif de taux réduit de TVA constitue une part très importante de l'aide de l'État à la production de logements sociaux. Pouvoir en bénéficier permet aux bailleurs de baisser le niveau de loyer de sortie des nouvelles opérations, mais aussi, à loyer égal, d'économiser sur leurs fonds propres afin de les réaffecter sur d'autres opérations. Les demandeurs de logements sociaux sont aujourd'hui au nombre de 2 millions les ressources dont ils disposent baissent régulièrement, encore plus avec cette crise, justifiant ainsi la construction massive de logements à loyer très modéré. En cette période de crise sanitaire et de crise économique, la relance de l'économie passe par un investissement massif dans la construction et la rénovation de logements, secteur créateur d'emplois non délocalisables. Les logements neufs contribueront en outre à renforcer la cohésion sociale et territoriale, en améliorant le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles. Au vu des plafonds de ressources et des plafonds de loyers des logements financés en PLS, la nécessité de disposer de la TVA à taux réduit sur ce produit est moins marquée.

La loi de finances pour 2020 a prévu l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux constructions de logements locatifs sociaux financés en PLUS qui font l'objet d'une convention de renouvellement urbain. Notre amendement tend à étendre ce régime aux logements locatifs sociaux construits dans le cadre des conventions de rénovation urbaine, qui correspondent au premier programme national de rénovation urbaine, en cours de finalisation, mais pour lequel certaines constructions ou reconstructions de logements locatifs sociaux ne sont pas encore livrées. Il ne serait pas logique que ces constructions soient taxées à 10 % alors qu'elles s'inscrivent pleinement dans le cadre de la politique de renouvellement urbain.

pour toutes les opérations, y compris celles déjà engagées, mais non encore livrées, entraînant un surcoût non prévu. Dans ces conditions, il paraît juste de revenir au taux de 5,5 % pour les opérations non encore livrées au 1 décembre 2019, sachant que le coût de la mesure sera limité, puisque la majorité des conventions de rénovation urbaine sont arrivées à échéance. Nous estimons que le coût serait de l'ordre de 5 millions d'euros, pour environ 700 logements financés en PLUS et non encore achevés. L'amendement

si vous ne voulez pas que nous soyons confrontés à une chute historique du nombre de logements produits, il est plus que temps que le Gouvernement nous dise où il veut aller, et comment. La parole est à Mme Valérie Létard,

il y a urgence pour le logement social, urgence à accompagner les bailleurs sociaux, pas seulement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais partout.

À l'Assemblée nationale, le Gouvernement a rejeté un amendement similaire, qui était soutenu par le rapporteur général

Ces opérations permettent en effet la création de nouveaux logements sociaux à partir de la transformation d'immeubles anciens de bureaux ou de logements privés. La loi a retenu une définition stricte de ces opérations d'acquisition-amélioration, qui conduit à écarter certaines opérations qui, pourtant, correspondent

en vue de sa transformation en logements sociaux, sont effectués, non pas par l'organisme acquéreur, mais par le vendeur dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover. On rencontre régulièrement ce type de situations, notamment dans les zones tendues où les montages réalisés sur des immeubles anciens sont souvent complexes. Je précise que, dans les deux cas visés, l'opération aboutit bien à la création de nouveaux logements locatifs sociaux, et que les conditions d'application du taux de TVA à 5,5 % restent encadrées par les mêmes conditions

madame la ministre

faisant l'objet d'opérations de renouvellement urbain. Dans celui-ci, les opérations d'accession sociale à la propriété bénéficiaient d'un taux de TVA réduit de 5,5 %. Ce périmètre a été a été ultérieurement restreint à 300 mètres pour permettre des économies budgétaires et pour éviter de diluer les effets de la mesure, étant donné qu'il reste difficile de réaliser de telles opérations à l'intérieur même de ces quartiers. Cette mesure et ce périmètre méritent d'être revus au regard d'études récentes de l'Insee et de l'Institut Paris Région sur la ségrégation sociale et la mobilité des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. En effet, loin des stéréotypes souvent très négatifs, ces études nous laissent percevoir un visage différent de ces quartiers, qui ne sont pas des trappes à pauvreté, mais des lieux où une réelle mobilité et une ascension sociale sont possibles et doivent être encouragées. L'un des signes de cette ascension sociale est la mobilité résidentielle, le déménagement et, plus encore, l'accession à la propriété. Or qu'observe-t-on ? On constate que l'on déménage autant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville que dans le reste de l'Île-de-France, dans la moitié des cas, hors de la géographie prioritaire et que, dans un peu moins de la moitié des cas, le déménagement conduit à un changement de statut d'occupation, notamment vers la propriété.

de mixité et d'interpénétration entre le quartier et le reste de la zone urbaine environnante, qui vient conforter la réussite des programmes de rénovation urbaine : ceux-ci ont en effet pour but d'introduire une plus grande mixité d'habitats, de fonctions et de populations dans les quartiers eux-mêmes, mais aussi à leur périphérie pour les diluer dans la ville. Pour amplifier ces bons résultats

Toutefois, cette dernière condition n'est pas applicable dans les quartiers faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain ou dans les communes qui comportent 35 % de logements locatifs sociaux, afin de favoriser la mixité. L'amendement un double objet. D'abord, il tend à simplifier la procédure administrative, ce qui est assez rare pour être souligné ; ensuite, il vise à élargir le dispositif. En ce qui concerne la procédure administrative, nous proposons de remplacer le calcul du seuil afférent à cette clause dans le sens d'un assouplissement, en recourant à une proportion évaluée non plus en mètres carrés de logements, mais en nombre de logements, ce qui est plus simple.

l'investisseur institutionnel est usufruitier des logements mis en location, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Il est également étendu, afin de limiter les impacts sur l'artificialisation des sols, à l'ensemble des transformations de locaux qui ne sont pas à usage d'habitation, au-delà des seuls locaux à usage de bureaux.

de transformation en zone urbaine. Afin de promouvoir la production de logements intermédiaires par la transformation de locaux existants, nous proposons que ces logements puissent être construits, non seulement en remplacement de bureaux, mais aussi à travers des opérations de transformation portant sur tous types d'actifs. Cet amendement s'inscrit pleinement dans la volonté actuelle des acteurs publics de renforcer une culture de la reconversion de l'existant, à l'opposé des opérations de démolition-reconstruction plus coûteuses sur le plan environnemental et plus souvent contestées par les riverains. Or il arrive régulièrement que des opérations de réhabilitation véritablement exemplaires sur les plans architectural et environnemental se voient refuser l'octroi d'un agrément pour le logement locatif intermédiaire, car les locaux en question ne sont pas considérés juridiquement, à la lecture des textes, comme des bureaux. Il apparaît donc souhaitable de soutenir ce processus vertueux sur le plan environnemental en autorisant la réalisation de logements intermédiaires dans ces projets, qui pourront dès lors s'accompagner de la production de logements pour les classes moyennes.

et de plus de 15 milliards d'euros d'importations annuelles de pétrole et de gaz. Si les nouvelles constructions sont « énergétiquement » performantes, la majorité du parc immobilier, qui ne se renouvelle qu'au rythme de 0,1 % par an, est constituée de bâtiments dont le niveau de consommation reste élevé. Au-delà des considérations environnementales, la rénovation concerne aussi la sauvegarde du patrimoine bâti, la balance commerciale française et l'emploi. Pourtant, la rénovation thermique de l'existant est peu présente dans le cadre réglementaire et législatif français. Les rénovations thermiques spontanées sont rares : on estime à 10 000 par an, environ, le nombre de celles qui amènent le logement vers les classes A ou B2. Cet amendement vise à élargir le taux réduit de TVA à l'ensemble des travaux de rénovation énergétique sur les bâtiments publics, ainsi qu'à favoriser la réalisation de bouquets de travaux qu'il conviendra de définir par voie d'arrêté.

pour accroître la performance énergétique de leur patrimoine et, ainsi, de voir une baisse des charges supportées par les locataires du parc social. En effet, depuis 2018, et contrairement à ce qui a pu être indiqué à l'Assemblée nationale en première lecture, seule une liste restreinte de travaux de rénovation énergétique peut bénéficier du taux de 5,5 % en application de l'article 278-0 A du code général des impôts, les autres travaux étant taxés à 10 %. Le législateur a déjà pris en compte cette situation par le passé. Ainsi, entre 2014 et 2018, les bailleurs sociaux ont bénéficié du taux de 5,5 % sur l'ensemble de leurs travaux d'économie d'énergie, au-delà de la seule liste de travaux visés à l'article 278-0 A, avant que ce régime soit supprimé en 2018, entraînant un surcoût au titre de ces opérations de rénovation. La parole

madame la ministre

l'amendement ne renvoie à aucune exigence technique ou norme de qualité environnementale quant aux systèmes et équipements concernés ou aux qualifications des prestataires. au regard de l'objectif environnemental visé, il ne nous paraît pas logique de faire une différence entre secteur libre et secteur social. L'enjeu est de réduire les émissions de CO2, là où on peut le faire et le plus rapidement possible.

sous l'autorité de Bernard Cazeneuve, a bénéficié d'un accompagnement total et plein d'énergie du président de la région, des deux présidents de département et de huit présidents d'intercommunalité. C'est un enjeu énorme pour ce territoire ; c'est un espoir que nous pouvons redonner ses habitants qui vivent souvent dans des logements totalement inadaptés, de véritables épaves énergétiques. À l'époque florissante du bassin minier, on chauffait gratuitement au charbon.

un vote positif.

avec 3 300 réhabilitations de logements- cela représente une multiplication par deux du nombre de logements ayant vocation à être réhabilités chaque année

sur la création d'entreprises génératrices d'emplois sur le territoire. Voilà le cadre dans lequel nous intervenons. J'entends que l'on pourrait abaisser le taux de TVA ponctuellement pour accompagner telle ou telle politique publique. C'est le jeu du projet de loi de finances

situation et d'un patrimoine exceptionnels. Le bassin minier a chauffé la France. Il a permis la deuxième révolution industrielle. Aujourd'hui, il souffre.

D'ailleurs, le seuil de la franchise en base, spécifique à la profession d'avocat, est bien plus avantageux que le seuil de droit commun applicable aux prestations de services en général. Enfin, les avocats peuvent, en parallèle, bénéficier d'une franchise spécifique de 18 300 euros pour les activités autres que celles définies par la réglementation applicable à leur profession. Pour toutes ces raisons, il ne nous semble pas

voulons ainsi protéger les publics jeunes des publicités pour des produits, dont les taux en sel, en gras et en sucre ou l'ultra-transformation dépassent les recommandations nutritionnelles. Les fonds récoltés permettraient de financer la promotion d'une alimentation saine et durable. faudrait pas pénaliser les petites et moyennes entreprises ou les exploitants agricoles menant des actions de publicité à petite échelle : cette taxe concernerait donc uniquement les entreprises, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros.

n'est pas habilitée à distribuer le crédit d'impôt pour l'acquisition de charges pour véhicules électriques. C'est pourquoi l'article 12 proroge le crédit d'impôt destiné à l'acquisition et à la pose de systèmes de recharge pour de tels véhicules. Madame la ministre, l'examen de cet article de dire quelques mots du dispositif MaPrimeRénov'et, plus globalement, de la politique du Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments. C'est un enjeu de tout premier ordre : au niveau national, le secteur du bâtiment représente près de 25 % des émissions de gaz à effet de serre, dont environ les deux tiers sont issus du secteur résidentiel. À cet égard, la rénovation énergétique des logements est une opportunité majeure : ses bénéfices environnementaux, mais aussi économiques et donc sociaux

L'article 12 crée un nouveau crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour installer une borne de recharge électrique. Le montant du crédit d'impôt est porté à 75 % du montant des dépenses éligibles effectivement supportées, dans la limite de 300 euros par système de charge. tel équipement représente un coût significatif pour les ménages. Si l'on veut vraiment lever les freins actuels au développement du véhicule électrique en France, il convient notamment d'inciter les particuliers à s'emparer de ce dispositif, en le rendant plus efficace.

un avis favorable

les communes ne pouvant plus délibérer sur le montant du produit à percevoir, elles seront soumises à l'État. Madame la ministre, vous entendez que les communes soient gérées non par des élus, mais uniquement par des agents d'exécution,

on peut comprendre le souci de simplification et de regroupement de la gestion dans un guichet unique,

D'ici à 2023, les collectivités ne pourront plus délibérer sur le montant du produit à percevoir. En outre, quel sera l'impact pour les ménages d'une tarification locale de l'électricité portée au maximum ?

qui perçoivent cette taxe. Cet article prévoit, d'une part, la fusion des trois systèmes actuels de taxation, communal, départemental et national, d'autre part, le transfert de la gestion du recouvrement de cette taxe unifiée à la Si l'on ne peut que souscrire à la volonté de simplification à laquelle répond cet article, je me dois de relayer les craintes que suscitent les dispositifs proposés. En uniformisant le système de taxes pour ne retenir, d'ici à 2023, qu'un seul taux, l'article 13 porte une atteinte à la liberté,

comme pour la taxe d'habitation ? Par ailleurs, cette uniformisation impliquant un alignement sur le taux maximal, on peut craindre ses répercussions sur la facture d'électricité des consommateurs, particulièrement dans les communes où le taux est actuellement faible ou nul. Enfin, le système proposé substitue au versement de la taxe aux collectivités le versement d'une part communale or les collectivités souhaiteraient avoir l'assurance que ces reversements seront effectués de manière régulière et qu'ils tiendront compte des évolutions locales. Il s'agit, pour elles, d'obtenir la garantie que les montants les montants de taxe reversés à partir de 2023 correspondront bien aux quantités d'électricité délivrées sur leur territoire. Le Sénat représente les collectivités au plus près. C'est pourquoi je présenterai des amendements visant à apaiser ces craintes. l'article. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, quelques mots sur cet article 13

entre les collectivités du bloc communal et les départements, conformément à la loi de décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, Globalement, le rendement annuel de cette taxe s'élève à 10 milliards d'euros, dont 7,7 milliards pour la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité 2,3 milliards de taxes communales et départementales. S'agissant de la taxe communale, la compétence est essentiellement allouée à des groupements de communes et je tiens à mentionner l'importance du rôle de proximité des syndicats intercommunaux et des fédérations de l'énergie qui, au fil des années, ont réalisé beaucoup de travaux sur

d'électricité (TCCFE), un prélèvement réalisé par les fournisseurs d'électricité sur les factures, dont le produit est ensuite reversé aux communes au titre de l'exercice de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité.

Le Gouvernement avait indiqué qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôt, mais l'article 13 porte une hausse de l'imposition pour les habitants des communes qui appliquaient jusqu'ici un taux zéro. zéro. Il aura des conséquences négatives sur le pouvoir d'achat des Français, tout en affaiblissant une nouvelle fois le pouvoir des collectivités et de leurs groupements

européennes, de faire perdre aux taxes locales sur la consommation finale d'électricité leur caractère local. Ces taxes seraient englobées dans une taxe nationale unique, réservée par quote-part aux bénéficiaires locaux. S'il est, comme toujours, présenté sous couvert de simplification et d'harmonisation,

s'agit de taxes pour lesquelles les collectivités disposent encore d'un pouvoir de taux, ce qui est de plus en plus rare. Cette taxe sur la consommation finale d'électricité est importante : elle représente 2,3 milliards d'euros, dont 906 millions d'euros pour le seul bloc communal. en outre, que cette petite marge de manoeuvre laissée aux collectivités, même très encadrée, leur permettait d'agir pour la transition écologique en dehors des politiques centralisées. Le Gouvernement parle à tout va de territorialisation des politiques, mais introduit de telles mesures qui reviennent à imposer une recentralisation très forte. Au-delà des questions relatives à l'autonomie fiscale locale,

les taux sont faibles. Au final, l'augmentation risque de ne pas être anodine.

4 euros et 30 euros dans 6,6 % des communes et entre 10 euros et 55 euros dans 5,2 % des communes. Ainsi, l'intégration des deux taxes locales au sein de l'actuelle TICFE entraînera entraînera un recul du pouvoir fiscal des collectivités territoriales et une hausse de la pression fiscale résultant de l'alignement progressif des coefficients multiplicateurs- cette hausse ne doit pas être négligée.

la balle est dans le camp du Gouvernement, lequel dispose d'un mécanisme d'accompagnement des ménages les plus précaires, le chèque énergie, dont le taux de recours est encore

20 % des communes et, jusqu'à preuve du contraire, cela ne fait pas 20 % des habitants ! Je ne vais pas vous expliquer la différence entre une commune de 100 habitants et une commune de 2 millions d'habitants, vous la connaissez mieux que moi. Il ne s'agit évidemment pas de

sont livrées à un consommateur, mais que ce dernier ne règle pas sa facture. En l'état actuel du droit, le fournisseur est tenu d'acquitter la taxe, dès lors

la Convention citoyenne pour le climat proposait deux ans. Ce lissage sur trois ans que vous proposez, madame la ministre, est un exemple parmi d'autres de votre manque d'ambition. est l'outil de référence pour mettre en oeuvre des mesures environnementales à la hauteur des enjeux climatiques et pour répondre à la demande populaire, de plus en plus grande en la matière. Malheureusement, madame la ministre, bien aidée par nos collègues de la majorité sénatoriale, vous ne faites les choses qu'à moitié Vous avez édulcoré au maximum les mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Comment allez-vous réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d'ici à 2030, avec des mesures si timorées ? l'article 14 est le symbole de la timidité, voire de la duplicité, du Gouvernement sur les questions environnementales : beaucoup de tapage médiatique sur la Convention citoyenne pour le climat, mais, dans les faits, c'est une autre musique que nous chante le Gouvernement les amendements portant baisse de la TVA à 5,5 % pour les mobilités collectives du quotidien ont été rejetés, de même que la réforme de l'indemnité kilométrique dans le barème de l'impôt sur le revenu, qui avantage aujourd'hui les voitures puissantes. est donc une nouvelle occasion manquée par le Gouvernement. Madame la ministre, soyez ambitieuse ! La question environnementale ne doit pas passer au second plan

la même exonération de taxe annuelle sur les véhicules de société en 2021 et de taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone à compter de 2022

au superéthanol E85, en dessous d'un certain seuil d'émissions.

a pour objet d'accorder, à partir du 1 janvier 2022, une exonération de taxe sur les véhicules de société de trois ans aux véhicules fonctionnant, depuis l'origine, au superéthanol E85, en dessous d'un certain seuil d'émissions.

Aligner le régime d'abattement applicable au calcul de la TVS sur celui de la prime à la conversion et du malus pour les véhicules « flexfuel » E85 d'origine est une mesure de neutralité technologique, de cohérence et d'égalité devant l'impôt, puisqu'il s'agit d'harmoniser les règles

l'électricité ou l'hydrogène avec le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85, soit

que vous éclairiez notre assemblée et le rapporteur général que je suis sur les raisons qui ont conduit le Gouvernement à ne pas faire bénéficier de cette exonération les véhicules utilisant le mélange essence-superéthanol E85. Madame la ministre,

bénéficient également d'une exonération, sous réserve de respecter certains seuils. Ces divers avantages, qui ont été étendus l'année dernière, fonctionnent : les ventes de superéthanol E85 croissent fortement.

vote. Madame la ministre, je suis étonné de l'analyse que vous faites- c'est une vieille analyse

propose un lissage du barème de la taxe sur les véhicules de société. Cependant, ce nouveau barème ne prend pas en compte le poids

appliqués jusqu'au seuil de 1,7 tonne. Cela permettrait de favoriser la transition écologique du parc des véhicules de société, parc qui représente près de la moitié des achats de véhicules neufs. Quel est l'avis de la commission

la possibilité d'un calcul forfaitaire, sur une base trimestrielle, de la proportion annuelle d'utilisation d'un véhicule. Ce mode de calcul, qui n'existe pas aujourd'hui pour la taxe spéciale sur certains véhicules routiers et qui constitue le mode de calcul de droit commun pour la taxe sur les véhicules des sociétés, devient optionnel

Or ce mode de calcul n'existe pas aujourd'hui pour la taxe spéciale sur certains véhicules routiers. Il ne serait pas cohérent de l'introduire pour une année seulement, alors même que la gestion de cette taxe est profondément réformée en 2021 dans le cadre de son transfert à l'administration fiscale. En outre, s'agissant de la taxe sur les véhicules des sociétés, les entreprises ont exprimé le souhait de disposer d'un temps d'adaptation plus long. C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise

Rappelons qu'en 2020 le malus avait déjà connu le plus fort durcissement de son histoire, ses montants ayant augmenté dans toutes les tranches et pour toutes les gammes de véhicules, y compris les plus populaires. L'achat d'une Clio IV à essence ou d'une Peugeot 308 au gazole n'occasionnait aucun malus en 2020, mais donnerait lieu à un malus de 150 euros en 2021 et 310 euros en 2022. Un véhicule Peugeot 3008 à essence, assemblé à Sochaux, ne se voyait appliquer aucun malus en 2019, alors qu'il occasionne cette année un malus de 210 euros. Ce montant passerait à 360 euros en 2021 et à 983 euros en 2022. Une Scénic à essence, fabriquée à Douai, se voyait appliquer un malus de 90 euros en 2019, montant qui a été porté à 818 euros en 2020 et qui atteindrait 1 504 euros en 2021, puis 2 726 euros en 2022. Il convient de refuser ces nouvelles hausses de la taxation des achats de véhicules neufs ; elles ne sont pas les bons leviers de verdissement du parc automobile, mais simplement des mesures de rendement budgétaire. Nous déplorons cette logique d'une écologie purement punitive ; dans le cas présent, les recettes du malus perçues par l'État sont supérieures au montant total des bonus versés aux Français.

avant même qu'elle soit mise en place, une région de France s'est levée et la ministre de l'époque a retiré le dispositif. Vous savez ce qu'il en a coûté aux finances publiques ... Le deuxième exemple

vise à augmenter le barème du malus automobile assis sur les émissions de CO2. Il répond à la nécessité de saisir l'opportunité de la relance et du soutien offert à la filière automobile pour orienter le secteur vers des véhicules peu émetteurs et légers, compatibles avec l'ambition écologique du Gouvernement, et pour écarter le risque d'une relance opérée au détriment de la transition écologique.

de l'article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ? Avis

d'une réduction des impôts de production, je souhaiterais qu'il intègre le fait qu'un véhicule de société n'est ni un gadget ni un luxe ostentatoire, mais un outil de production

certain nombre de simplifications dans le cadre du transfert de la taxe à l'essieu de l'administration des douanes et des droits indirects à l'administration fiscale.

Cet amendement vise à faire coïncider la réfaction au bénéfice des familles avec la nouvelle grille de malus, en l'augmentant de cinq grammes par enfant, soit quinze grammes pour trois enfants, ce qui équivaut à l'abaissement du seuil du malus.

que vous proposez me semble contraire à la finalité environnementale de la taxe, qui est assise sur les émissions de CO2 et pas sur l'endroit où l'on utilise le véhicule. Une émission de CO2 reste une émission de CO2

ou modifier ses pratiques. Seules les caractéristiques techniques du véhicule permettent d'asseoir une taxe de manière sécurisée pour le redevable comme pour les pouvoirs publics.

comme l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Certaines régions ont mis en place ce système qui permet de concilier écologie, pouvoir d'achat et accompagnement au passage à un véhicule propre. Il serait opportun de le déployer à l'échelle du pays. Sur le fond, le Gouvernement n'y semble pas totalement opposé, puisqu'il a donné un avis favorable à un amendement de notre collègue député Dino Cinieri, lequel a pour objet de réfléchir à un élargissement de cette exonération. Il me semble nécessaire d'aller plus vite et plus loin, plutôt que de passer par l'étape intermédiaire d'un énième rapport.

satisfait. L'exonération systématique des véhicules électriques à hydrogène est entrée en vigueur au 1 janvier 2020.

à M. Bernard Delcros. Cet amendement a été déposé par M. Hervé Marseille. Le malus automobile vise à taxer les véhicules en fonction de leurs émissions de CO2. Cependant, les véhicules à forte capacité d'occupation, qui comprennent plus de cinq places assises, permettent de diminuer l'empreinte écologique de chaque passager transporté. avec 12 % des immatriculations en France, les entreprises de location de courte durée ont un rôle à jouer dans la transition vers une mobilité plus propre et responsable. Elles apportent une solution alternative à la possession d'un véhicule et contribuent à la réduction de la pollution liée aux transports terrestres. Un véhicule partagé d'une société de location remplace huit véhicules individuels. Les loueurs de véhicules de courte durée favorisent le partage effectif d'un même véhicule entre de nombreux locataires et incitent les conducteurs à passer de la propriété à l'usage en fonction des besoins. Le présent amendement propose que les véhicules d'au moins cinq places assises, acquis par les entreprises de location de courte durée, bénéficient d'une réfaction de cinquante grammes sur les émissions de CO2 pour le calcul de leur malus. Il s'agit, en réalité, d'une mesure favorable à l'environnement.

Le système de bonus-malus automobile favorise le choix d'un véhicule peu émetteur de CO2 et pénalise l'achat des modèles les plus polluants. Cependant, les véhicules à forte capacité d'occupation comprenant sept places assises permettent également de diminuer l'empreinte écologique de chaque passager. Au-delà de la contribution à la réduction de la congestion et du nombre de véhicules sur la route, ces véhicules remplissent aussi un rôle social. Avec 12 % des immatriculations, les entreprises de location de courte durée jouent un rôle majeur dans la transition vers une mobilité plus propre et responsable. Elles apportent une solution alternative à la détention individuelle d'un véhicule. En effet, pour le transport de petits groupes, la réduction du malus pourrait devenir incitative et permettre l'essor d'un transport groupé plus vertueux.

assises, acquis par des personnes morales, est prévu à l'alinéa 200 de l'article 14 du présent PLF. À l'image de ce dispositif, le présent amendement propose que les véhicules de sept places assises, acquis par les entreprises de location de véhicules de courte durée, bénéficient d'une réfaction de cinquante grammes sur les émissions de CO2 pour le calcul de leur malus. Quel

émissions. Il a pour objet de relever le barème d'amortissement déductible de l'impôt sur les sociétés, en le faisant passer de 30 000 euros à 40 000 euros pour les véhicules à très faibles émissions et de 20 300 euros à 25 000 euros pour les véhicules à faibles émissions.

une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Il s'agit de moduler le remboursement des frais de déplacement déductibles de l'impôt sur le revenu en fonction des émissions de CO2 et du poids des véhicules.

Par ailleurs, la Cour des comptes, dans un rapport de 2020 sur les politiques de lutte contre la pollution de l'air, suggérait, elle aussi, de prendre en compte le poids dans la fiscalité des véhicules. Enfin, le renforcement du barème du malus automobile est complémentaire de la création d'une fiscalité assise sur le poids des véhicules. Ces deux mesures sont nécessaires pour restaurer l'efficacité des outils français de décarbonation du parc automobile.

une vision, de la lisibilité pour amener progressivement les Français à adhérer à la démarche. Vous le savez, puisque nous avons souvent partagé le même point de vue, sans être de même conviction, ce n'est pas l'addition de taxes, jusqu'au moment où elles finissent

en envoyant un signal clair aux donneurs d'ordre, c'est-à-dire aux responsables du choix des transports. Autrement dit, c'est un principe d'écotaxe qui s'appliquerait non pas aux transporteurs, mais à ceux qui commandent les transports, les donneurs d'ordre. Ce dispositif est pragmatique, puisqu'il est fondé sur un dispositif

à cet endroit de la chaîne un système de taxation pour avoir un dispositif pollueur-payeur très pédagogique et vertueux.

principalement destiné à l'écoute de musique afin de corriger une anomalie, puisque ce secteur bénéficie de la création, sans la financer. Il s'agit d'un marché dynamique, principalement porté par des entreprises extraeuropéennes, qui représente 20 millions d'unités vendues. taxe est suffisamment large pour nous permettre d'appliquer un taux très faible, 1 %, afin de minimiser tout risque de répercussion sur le consommateur. Il est également proposé de ne pas affecter cette taxe pour permettre au Gouvernement de soutenir d'autres acteurs du monde sonore que le CNM, par exemple

aujourd'hui des vecteurs importants de consommation musicale. La combinaison de ces deux éléments fait de cette taxe une TVA qui s'appliquerait de façon arbitraire à certains matériels d'écoute et en exonérerait d'autres. C'est la raison pour laquelle je sollicite le retrait de ces amendements. ? Je vais reprendre les arguments de M. le rapporteur général. L'avis est défavorable, d'abord parce que c'est une nouvelle taxe

ainsi libellé : La parole est à M. Patrice Joly. Cet amendement vise à créer une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l'achat de véhicules polluants, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone dépasse 95 grammes par kilomètre.

dépensent chaque année 34 milliards d'euros, tous supports confondus, à la publicité pour les véhicules, donc pour des produits polluants. Cette taxation représenterait un levier puissant qui devrait, selon nous, être mis au service de la transition énergétique et de la sobriété dans l'utilisation des ressources- ces sommes pourraient par exemple être fléchées vers le développement des transports collectifs. Quel

En l'absence d'informations relatives notamment à la composition de l'activité, à l'évolution des prix ou à l'emploi, le Haut Conseil ne dispose pas de l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de toute prévision macroéconomique et plus particulièrement à celle des principaux déterminants des recettes publiques. souligne que le Gouvernement, sur la base de la rédaction de l'article 16 de la loi organique de 2012, qui prête à interprétation, a choisi de retenir une lecture étroite de ce texte, en ne présentant pas au Haut Conseil de nouvelles prévisions de finances publiques- recettes, dépenses et soldes.

le Haut Conseil a endossé les prévisions de croissance, sur lesquelles nous allons asseoir le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il a qualifié notre prévision 2020 de prudente et la croissance 2021 de cohérente avec les hypothèses sanitaires que nous avons choisies. Nous allons maintenant tirer les conséquences des révisions macroéconomiques sur les textes financiers pour l'année 2021.

Je crois que l'on peut souligner, et je sais que vous en êtes conscient, que nous sommes dans une situation d'incertitude extraordinaire, au regard non seulement de la situation sanitaire, mais aussi de paramètres comme le Brexitou

d'assurance automobile, dont le tarif pourrait être fonction, notamment, des émissions de gaz à effet de serre. Le poids moyen des voitures neuves a beaucoup augmenté ces dernières années, notamment en raison de la hausse des ventes de SUV. Ces derniers comptent aujourd'hui pour près d'un tiers du marché européen ; prendre en compte le poids des véhicules dans le calcul du bonus-malus écologique paraît donc essentiel pour répondre aux défis actuels et intégrer les évolutions de la demande et des comportements. Quel est l'avis de la

je vous le dis, elle devient complètement illisible. Ensuite, le dispositif proposé ne me paraît pas pertinent, parce qu'il s'ajoute à d'autres taxes similaires, dont

(TSCA), pendant trois ans, les contrats d'assurance des véhicules électriques immatriculés à compter du 1 janvier 2021. Vous le voyez, le choix que nous faisons est de faciliter la transition vers les voitures électriques. Il ne s'agit pas de taxer davantage des gens qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule.

bonus et de malus écologiques à l'achat sont fondés, notamment, sur la valeur des émissions de CO2. La prise en compte de la valeur unitaire des émissions nécessite la transmission des données du certificat de conformité du véhicule en format électronique.

constituent un instrument économique équitable et efficace pour réaliser une politique des transports durable, puisqu'ils sont directement liés à l'utilisation de l'infrastructure. » La redevance kilométrique existe déjà dans certains pays comme l'Allemagne, l'Autriche ou la Belgique. Contrairement au système de la vignette, la redevance kilométrique tient compte du nombre de kilomètres parcourus par les transporteurs. Il s'agit d'appliquer le principe du pollueur-payeur. Le montant de cette taxe serait progressif afin de limiter, à moyen terme du moins, l'emploi du transport routier sur de longues distances, dans la mesure où il présente un bilan carbone très problématique. Une telle mesure permettrait de réduire la demande et, incidemment, d'optimiser le transport routier de marchandises, en favorisant d'autres modes de transports. Un amendement à l'objet identique avait déjà été déposé par le groupe socialiste du Sénat à l'occasion de l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités. Un tel dispositif s'inscrit parfaitement dans la lignée des propositions de la Convention citoyenne pour le climat.

La fiscalité actuelle retient déjà la logique du principe utilisateur-payeur et fait participer les transporteurs au financement des infrastructures. 2015, l'augmentation de 4 euros par hectolitre de l'accise sur le gazole professionnel pour le transport de marchandises a été privilégiée. De plus, pour couvrir la programmation des infrastructures prévue dans la loi d'orientation des mobilités, il a été décidé que le transport routier de marchandises contribuerait sous la forme d'une nouvelle diminution du remboursement partiel de la TICPE à hauteur de 2 euros par hectolitre

à la frontière espagnole avec un plein de carburant acheté dans le Grand-Duché. Nous avions donc adopté un système qui était pertinent

Rotterdam est le plus grand port méditerranéen ! -, vous observez un flux de poids lourds que vous ne maîtrisez pas et qui s'impose à vos infrastructures sans leur apporter aucune contribution.

Si Mme Royal avait eu la patience d'ouvrir une négociation avec les régions pour différencier le taux de prélèvement, peut-être aurait-elle tout de même affronté crises et critiques, mais un système qui a somme toute coûté au contribuable français plus d'un milliard d'euros et ne nous laisse pour tout souvenir que des portiques aurait pu commencer à fonctionner. Alors, soyons sérieux : votre démarche est bonne,

en charge facultative par les employeurs des frais de déplacement de leurs employés par les transports en commun ou les nouvelles mobilités- abonnement de covoiturage, vélo, engins de déplacement personnel. Ce forfait est exonéré d'impôt sur le revenu et de cotisations

l'avis de la commission ? J'ai le sentiment que les entreprises qui choisiraient d'offrir à leurs salariés le cumul du forfait mobilités durables et du remboursement partiel des frais de transports en commun

est louable. Néanmoins, un blocage subsiste pour l'efficacité du dispositif, puisque ce plafond reste encore trop bas pour permettre la prise en charge totale par l'employeur des frais de déplacement de ses salariés et assurer ainsi une politique intermodale favorable aux transports collectifs et à la mobilité douce. Mes chers collègues, j'en appelle à votre bon sens : il est normal qu'un dispositif mis en place si récemment ne soit pas parfait et nécessite des ajustements. Il faut l'améliorer ! L'adoption de cet amendement permettrait de corriger un obstacle à la bonne mise en oeuvre du forfait mobilités durables,

en portant de 400 euros à 500 euros l'exonération de cotisations sociales applicable à la prise en charge par l'employeur des frais engagés par les salariés pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail. Le présent amendement vise à relever également, dans ce cadre, la limite d'exonération pour la prise en charge par l'employeur des frais de carburant, en la portant de 200 euros à 300 euros. En effet, ce seuil instauré en 2008 n'a jamais fait l'objet d'une réévaluation malgré l'inflation et la hausse des prix du carburant. Au regard de la crise actuelle, privilégier une exonération destinée aux seuls véhicules propres serait discriminant pour les salariés qui n'ont pas la capacité financière d'y accéder ; cela a été démontré à plusieurs reprises, en particulier par Mme Lavarde

Nous vous proposons un allégement de cette taxe, en raison de son caractère particulièrement élevé pour une activité

Le montant à payer peut rapidement s'avérer prohibitif, ce qui constitue un frein à la préservation de certains véhicules, dont l'ancienneté est assortie de caractéristiques techniques qui justifient leur préservation. proposons aurait un impact tout à fait négligeable sur le budget de l'État, puisque, sur les vingt dernières années, moins de 10 000 véhicules, tous types, catégories et cylindrées confondus, sont immatriculés en moyenne chaque année en France dans la catégorie des véhicules de collection,

Aussi, le plafonnement à vingt chevaux fiscaux de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules de collection assurant les reconstitutions et commémorations historiques apparaît constituer une mesure de nature à renforcer la bonne préservation de notre patrimoine automobile historique. Très bien ! Quel est

sont un hommage rendu au travail de l'industrie française et étrangère, mais aussi une leçon d'espérance : si nous avons pu passer de véhicules bruyants, dangereux et incertains dans leur conduite et leur tenue de route à des voitures plus fiables qui ont largement contribué à la diminution du nombre de morts sur les routes, c'est bien grâce à cette évolution ! De la même façon que l'on apprend l'histoire de son pays, il me paraît utile de conserver l'histoire de notre patrimoine mécanique ! La parole est

Longuet l'a dit, c'est rendre hommage à ceux qui les ont construites ; c'est aussi rendre hommage à ceux qui les ont conduites, à ceux qui ont traversé la Manche avec leurs Jeeps ou leurs Dodge

Bien que ce dispositif constitue une avancée notable, il reste facultatif. La mise en place de dispositifs en faveur des mobilités douces a démontré que leur caractère facultatif n'est pas suffisant pour assurer leur mise en oeuvre. L'indemnité kilométrique vélo en est une illustration parfaite : à ce jour, 237 000 salariés, bénéficieraient de l'IKV. Répondons à la menace du changement climatique en permettant à l'ensemble de nos concitoyens de bénéficier de l'intermodalité pour leurs déplacements domicile-travail !

d'acides gras, afin de bénéficier,, de la taxation avantageuse déjà existante pour les biocarburants de type B100, à base de végétaux. Unique en Europe, cette innovation permettrait de répondre en partie aux demandes du Gouvernement, notamment celle de contribuer à la transition écologique

pour 2030. Il est important de rappeler que cette mesure permettrait d'atteindre plus de huit fois les objectifs européens énoncés. À l'heure actuelle, il n'existe pas d'autre solution permettant d'y répondre que celle ici proposée : une utilisation immédiate de cette innovation permettrait, dès à présent, une réduction d'un quart des émissions de gaz à effet de serre en flottes captives. Par conséquent, il serait souhaitable d'obtenir un allégement de TICPE, dès 30 % d'incorporation d'esters méthyliques d'acides gras applicables aux biocarburants avancés, du niveau d'incorporation. La

la commission ? Depuis le 1 janvier de cette année, les taux réduits de TICPE pour les produits équivalents au gazole ne sont plus conformes à la directive restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Le présent amendement a pour objet de maintenir à 0,4 % les seuils d'incorporation des égouts pauvres issus des plantes sucrières,

Les précédentes lois de finances avaient déjà introduit des augmentations de ce taux à 0,2 % en 2019, à 0,4 % en 2020 et à 0,8 % en 2021. Il est proposé de maintenir, à compter de 2021, le taux actuel de 0,4 %, afin de préserver les valorisations alimentaires de ces coproduits sucriers, lesquels constituent une matière première non substituable et particulièrement importante dans l'industrie de la levure. Une nouvelle augmentation de ces seuils d'incorporation ferait peser d'importants risques sur les approvisionnements des entreprises de ce secteur et pénaliserait fortement le développement des usages traditionnels et innovants des levures, pour le pain, le vin et la bière notamment. La filière est en effet engagée, sur le sol français, au développement de solutions d'avenir, telles que les produits de biocontrôle et biofertilisants pour diminuer l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques, probiotiques pour réduire l'usage d'antibiotiques dans les élevages et les protéines non animales pour une alimentation moins carnée ; autant de solutions s'inscrivant dans les objectifs du européen et du pacte productif qu'il convient d'encourager en permettant à la filière de sécuriser ses approvisionnements sur le territoire national.

Je ne suis pas favorable à des hausses supplémentaires du pourcentage cible d'incorporation d'énergies renouvelables dans les essences, qui risquerait de se traduire par une augmentation de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants acquittée par les redevables. Le taux d'incorporation de biocarburants dans les carburants fossiles doit, selon moi, augmenter régulièrement,

l'augmentation du taux d'incorporation et être attentif aux impacts sur le marché alimentaire du dispositif que nous sommes en train de construire sur les biocarburants.

progressivement. Cet amendement vise à conditionner l'extension de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants au secteur aérien à une étude d'impact sur les conséquences de l'augmentation de la demande en biocarburants avancés sur ce marché. à reporter l'extension prévue par le PLF, le temps de finaliser l'étude qui permettrait notamment d'évaluer l'adéquation entre les gisements disponibles en France et les usages envisagés. Il y a des biocarburants dits « propres » qui ne sont pas si propres que cela en réalité ! L'objectif d'augmenter la part de biocarburants dans le secteur aérien entraîne un fort risque d'importation de biocarburants contribuant à la déforestation. Les volumes de carburant nécessaires à l'aérien sont en effet importants alors que la production française de biocarburants avancés est limitée. Il convient donc

usagées importées, qui sont en réalité des huiles de palme ou de soja brut. La Chine, par exemple, exporte des volumes importants d'huiles alimentaires usagées vers l'Europe et importe, en substitution, de l'huile de palme, qui revient moins cher. C'est pour limiter ces risques que la directive européenne RED II a souhaité isoler ce type de biocarburants et fixer un seuil limite d'incorporation à 1,7 % dans les carburants routiers. En France, le gisement d'huiles alimentaires usagées est évalué à environ 100 000 tonnes par an. Selon les chiffres de l'Ademe, ce gisement est déjà valorisé à hauteur de 45 000 tonnes. Dans ce contexte particulièrement flou, la prudence commande de réaliser une réelle étude d'impact avant de se fixer un tel objectif pour le secteur aérien.

souhaitent, si je comprends bien, réduire les objectifs d'incorporation de biocarburants pour le secteur aérien, craignant que la filière française ne soit

une part de leurs craintes. Je considère qu'il nous faudra, le cas échéant, repousser l'entrée en vigueur de la Tirib au secteur aérien si la filière française de l'approvisionnement ne parvient pas à se structurer suffisamment avant le 1 janvier 2022. Pour tout vous dire, monsieur Labbé, des grandes

besoins. Je pense que l'on peut se dire les choses, dans le respect des sensibilités et des convictions de chacun. C'est la raison pour laquelle je demande le retrait